autour des enjeux suivants : agir pour une transition juste ; transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone ; s'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie ; agir pour la santé et le bien-être de tous ; rendre effective la participation citoyenne ; oeuvrer en ce sens sur les plans européen et international. Cette mesure donnerait aux producteurs de biens et de services la possibilité de valoriser leurs produits et d'informer parfaitement les consommateurs sur leur bilan en la matière. Quel est l'avis de la commission ? Pour des raisons déjà évoquées, je ne suis pas favorable à ce que nous complétions la rédaction de l'alinéa 4. Celui-ci doit rester simple pour être facilement compréhensible en vue du déploiement, sur le terrain,

Nous estimons que cette méthode de transparence peut s'avérer utile et qu'elle doit même être étendue, notamment aux produits financiers. En souscrivant un contrat d'épargne ou d'assurance, les citoyens financent l'économie aujourd'hui, il devient urgent de faire toute la lumière sur ce que l'on finance avec notre épargne. Si l'on ne souhaite pas financer des investissements dans les énergies fossiles ou des projets destructeurs de la biodiversité, il est important de pouvoir faire ce choix en toute transparence. Il semble donc nécessaire que les souscripteurs de placements soient pleinement informés de leurs choix en la matière, et ce d'autant plus que les sommes en question sont loin d'être négligeables ; l'encours des placements financiers des assureurs, par exemple, s'élève en France, en 2020, à plus de 2 700 milliards d'euros. Il paraît indispensable de connaître l'impact carbone Cet amendement s'inscrit dans un mouvement de fond visant au désinvestissement des banques des projets liés aux énergies fossiles. Récemment, le gouvernement néo-zélandais a présenté une loi obligeant les établissements financiers à évaluer l'impact de leurs activités sur le climat. Ne restons pas à la traîne ; la France doit, elle aussi, promouvoir une telle transparence en matière financière. Que les choix des citoyens-consommateurs

Or la possibilité, pour les professionnels, de recourir à la dématérialisation de l'affichage de l'impact environnemental est essentielle pour diverses raisons. L'affichage physique donnera lieu à une multiplication des supports d'information sur les produits et à une augmentation de leur taille, notamment pour ce qui est des petits produits.

Il s'agit de rendre cet affichage le plus universel possible, car, même si la très grande majorité des Français dispose aujourd'hui d'un smartphone, nous savons également que la maîtrise de son utilisation est pour le moins très inégale.

Nous craignons que l'inscription de cette exception dans la loi engendre des dérives et soit la porte ouverte à toutes les dérogations possibles et imaginables, rendant en conséquence le dispositif très opaque. Le présent amendement vise donc à prévoir que l'affichage environnemental devra se faire par voie de marquage ou d'étiquetage.

Quel est l'avis du Gouvernement ? nous sommes plutôt favorables à ne pas trop contraindre les choses dans la loi. Le décret permettra ensuite de définir les situations dans lesquelles il est plus adapté de choisir un étiquetage physique ou un étiquetage électronique.

ou du service mis sur le marché de détailler l'évaluation environnementale justifiant l'affichage retenu. En effet, l'affichage environnemental, quelle que soit sa forme, ne donnera que

Mme la rapporteure.

L'une ne peut fonctionner sans l'autre, notamment pour des raisons de transparence de l'information. Prenons l'exemple du commerce en ligne : le texte, en l'état, permettrait à la plateforme d'achat de choisir entre un affichage visible et un affichage accessible un lien plus ou moins évident pour l'acheteur.

il convient de ne pas contraindre davantage le cadre législatif. Les modalités d'affichage pourront être définies par voie réglementaire, sur le fondement des enseignements tirés des expérimentations qui sont en cours et en fonction des particularités de chaque secteur. Avis défavorable.

au travers de cet amendement, que l'affichage environnemental reste consultable par voie numérique après l'acte d'achat. Il s'agit de permettre la valorisation des produits de qualité. En effet, si cet affichage se fait par voie d'étiquetage

de valoriser les produits de qualité respectueux de l'environnement. Il paraît donc nécessaire que le consommateur puisse continuer d'avoir accès à cet affichage une fois passé l'acte d'achat. Quel est l'avis de la commission ?

consubstantielle d'une quantification de celui-ci et, d'autre part, en établissant une priorité entre certaines informations relatives aux impacts environnementaux. Cette priorité existe, mais il est proposé

essentielles, donc une dilution de l'intelligibilité. Il s'agit, en l'occurrence, de données à propos desquelles les consommateurs sont particulièrement sensibilisés depuis de nombreuses années. L'idée de hiérarchiser les informations relatives aux impacts environnementaux ne me semble pas aller dans le bon sens. Il faut garder de la souplesse et retenir la rédaction la plus claire et la plus épurée possible.

? Madame la sénatrice, votre amendement vise à ce que l'affichage fasse ressortir les impacts environnementaux de façon quantifiée et en tenant compte « principalement » des impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre

Cet amendement de précision vise à garantir au consommateur une information claire et synthétique sur l'impact environnemental des biens et services qui feront l'objet d'un affichage environnemental en application du présent article. Il tend également à préciser qu'il sera tenu compte, dans cette information agrégée, des impacts environnementaux les plus pertinents pour une catégorie donnée. Ces impacts environnementaux seront définis en concertation avec les parties prenantes des secteurs concernés.

que seul un affichage prenant en compte les dimensions environnementale et sociale répondra aux attentes de nos concitoyens d'une consommation plus juste et plus durable.

la rédaction actuelle revient à imposer ces trois éléments comme bases de l'affichage environnemental. Or l'objet même des expérimentations sera de déterminer quels sont les impacts les plus pertinents pour chaque secteur économique, afin d'adapter l'affichage à leurs particularités. Par exemple, concernant les produits textiles, l'affichage environnemental repose actuellement sur deux impacts : l'émission de gaz à effet de serre et l'eutrophisation de l'eau. Il convient donc de modifier la rédaction de cette phrase afin d'autoriser l'adaptation de cet affichage selon les secteurs.

Encore une fois, ce sont les expérimentations, auxquelles seront associées les parties prenantes, qui permettront de définir les modalités d'affichage pour une catégorie de produits donnés, y compris dans le cas où des critères sociaux sont pris en compte.

Cet amendement vise à ajouter une information sur le mode et le coût de transport d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services qui sont visés par l'article 15 de la loi du 10 février 2020, Les informations relatives au mode de transport et au coût de celui-ci sont devenues quasi inexistantes. Bien souvent, lorsqu'un consommateur passe une commande en ligne, il voit s'afficher « 0 euro » sur la ligne « Frais de port tout simplement parce que la distribution et les plateformes ont décidé, dans leur grande majorité, de faire passer ce service comme « gratuit » en l'imputant d'une autre manière dans le coût global d'un bien ou d'un service. Alors que la mondialisation à outrance des échanges a démontré ses limites en termes tant de développement durable et de préservation de notre environnement que de modèle social, l'information des consommateurs sur le coût et le mode de transport d'un bien ou d'un service constituerait un indicateur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et le combat pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement vise à informer les consommateurs de l'impact climatique lié au transport et à la livraison des produits. Si le fait de sensibiliser les consommateurs à l'empreinte carbone des produits constitue un progrès, rendre visible le coût carbone du transport permettra de responsabiliser l'ensemble des acteurs et incitera tant les consommateurs que les que les vendeurs à privilégier, au maximum, le recours aux transports décarbonés dans les chaînes logistiques, conformément aux objectifs de la Convention citoyenne pour le climat. Quel est l'avis de la commission ? Ces deux amendements

Un poulet brésilien transporté par voie de mer sur un porte-conteneurs de 20 000 équivalents vingt pieds (EVP) aura un impact carbone et monétaire beaucoup plus faible qu'un animal d'élevage transformé et transporté du sud vers le nord de la France avec un véhicule utilitaire léger ancien,

des externalités environnementales des produits qu'ils consomment, et ce en fonction de leur valeur nutritionnelle.

En valorisant les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs, sur les écosystèmes, des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés, les PSE s'intègrent totalement dans cette logique. Il faut ainsi reconnaître et encourager, en les rémunérant dans la durée, les éléments de biodiversité et les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique,

rectifié et 1068 rectifié tendent à introduire un critère nutritionnel dans l'affichage environnemental pour les produits alimentaires, ce qui n'a pas de lien, même indirect, avec le texte de cet article.

je ne suis pas favorable à cette proposition, qui conduirait à complexifier la mise en oeuvre de l'affichage environnemental, en faisant intervenir une nouvelle dimension économique. Toutefois, cette rédaction me semble bien

d'une mission spécifique sur l'affichage social ; je l'ai mentionné tout à l'heure. Cette plateforme fera des propositions sur la nature des indicateurs sociaux qui pourront être pris en compte dans le cadre du présent article. Il me semble toutefois préférable que les impacts considérés soient précisés dans les méthodologies et non dans la loi,

La lutte contre le réchauffement climatique doit s'accompagner d'une prise de conscience sociale sur les conditions de travail de ceux qui fabriquent les biens que nous importons. Nous l'avons rappelé, pour répondre à une véritable attente sociétale en matière d'environnement et de justice sociale, l'affichage environnemental ne peut faire l'économie de la prise en compte des critères sociaux. Cet amendement tend ainsi à prévoir que l'affichage atteste du respect des droits humains, notamment des droits des femmes et de l'enfant, sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

apportées aux consommateurs. Il y a donc un sujet de difficulté d'application. La multiplication des mentions sur les produits n'est pas souhaitable : l'information environnementale ou environnementale et sociale doit rester facilement lisible et accessible pour les consommateurs. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut,

La production agricole est au carrefour de nombreux enjeux. Parmi ceux-ci, le bien-être animal est une attente sociétale forte, souvent liée à l'environnement. C'est aussi pour de nombreuses productions, notamment pour la production bovine et laitière, un atout de nos filières locales. Dans toutes les productions animales agricoles, des méthodes de calcul non adaptées pourraient permettre à des produits importés d'avoir un meilleur score que des produits français respectant des normes de bien-être animal et environnementales supérieures. Comme le soulignait notamment l'interprofession bovine, les travaux sur l'affichage environnemental des produits alimentaires ont, pour l'instant, été plus que décevants, voire dangereux, pour notre élevage. Le dispositif Agribalyse, en s'appuyant sur l'analyse du cycle de vie et en ramenant ainsi l'impact sur l'environnement au kilogramme de produit, favorisera mécaniquement les systèmes intensifs et hors sol. Cette analyse ne reflète pas la complexité des produits alimentaires et favorise les plus hauts rendements, ce qui amène à des comparaisons pour le moins hasardeuses.

et a un moindre rendement au kilogramme de viande produite pour une même surface utilisée. Ces méthodes de calcul inadaptées sont absolument inacceptables, tant pour le producteur que pour le consommateur, car elles ne permettent pas

Cela permettra au système à l'herbe et au système bio d'être valorisés à la hauteur de leur impact réel. Cet amendement visait à compléter cette rédaction en insérant, dans l'affichage environnemental des produits issus de l'élevage, la prise en compte du bien-être animal, au même titre que les externalités

est à Mme Catherine Dumas. L'article 1 du projet de loi détaille les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir, le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage de l'impact environnemental L'article 15 de la loi du 10 février 2020 subordonnait le caractère obligatoire d'un affichage à « l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne poursuivant le même objectif ». Cette condition n'apparaît pas dans la nouvelle rédaction proposée. Or il est essentiel de prendre en compte les travaux que mène actuellement l'Union européenne sur le sujet de l'information du consommateur, avec le projet d'empreinte environnementale des produits. Depuis 2013, le projet européen a eu pour objectif d'élaborer des méthodes de calcul de l'impact environnemental des produits et services, et de tester des outils de communication auprès des partenaires commerciaux et des consommateurs. Le projet devrait prendre fin en 2023 et déboucher sur des propositions politiques de la part de l'Union européenne. Dans un souci de cohérence juridique au sein du marché unique européen, dans lequel s'inscrivent toutes les entreprises françaises, ainsi que dans un esprit d'égalité entre les producteurs français et leurs concurrents étrangers,

Il existe encore, à ce jour, trop d'incertitudes sur les méthodes d'évaluation environnementale pour préjuger les résultats des expérimentations, même si les travaux ont bien avancé. Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article 1 apporte déjà suffisamment de garanties sur le fait

S'il est utile que la France prenne de l'avance tant qu'une méthodologie commune n'est pas arrêtée, il sera nécessaire de respecter celle-ci une fois qu'elle sera définie. Ainsi, afin de limiter les risques de distorsion de concurrence due à la non-harmonisation des critères selon lesquels sont comparés les produits qui circulent au sein du marché unique, le présent amendement vise à inscrire clairement dans la loi que l'affichage environnemental ne peut être rendu obligatoire sans tenir compte des éventuelles dispositions de l'Union européenne visant le même objectif.

pour réellement orienter les consommateurs dans leur acte d'achat. Les évaluations qui seront conduites au terme des expérimentations permettront également d'analyser les enjeux économiques de cet affichage et de conclure quant à l'intérêt de le rendre obligatoire dans certains secteurs. L'objet de cet amendement est de ne pas préjuger les conclusions de ces expérimentations et de laisser les évaluations valider ou non le caractère obligatoire de l'affichage dans certains secteurs. L'amendement

L'industrie textile est l'un des secteurs économiques mondiaux qui, encore aujourd'hui, ont le plus recours au travail des enfants et au travail forcé. Les formes extrêmes de production qui se cachent derrière la mondialisation ont provoqué, au cours des dernières années, des catastrophes humaines désastreuses.

en témoignent les déplacements de milliers d'Ouïghours, organisés par l'État chinois dans les usines du territoire du Xinjiang, notamment pour la production de marques de textile telles qu'Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, Uniqlo ou H&M. Il est nécessaire de mettre fin à l'opacité qui entoure les conditions de travail des sous-traitants auxquels les multinationales de la mode ont recours lorsqu'elles cherchent à baisser le prix de leur main-d'oeuvre, voire lorsqu'elles organisent l'esclavage moderne. L'amendement n° 2107 à M. Frédéric Marchand. L'objet de cet amendement est de ne pas faire figurer le secteur alimentaire dans la liste des secteurs qui feront l'objet d'un affichage obligatoire. L'un des objectifs des expérimentations prévues au II de l'article 1 est précisément de déterminer les biens pour lesquels l'affichage sera rendu obligatoire. Il existe encore, à ce jour, trop d'incertitudes sur les méthodes d'évaluation environnementale pour préjuger les résultats des expérimentations, même si les travaux ont bien avancé. Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article 1 apporte déjà suffisamment de garanties sur le fait que l'affichage sera rendu obligatoire chaque fois qu'une méthode suffisamment robuste aura pu être conçue. Pour cette raison, il convient de prévoir que les expérimentations aient été menées à leur terme avant de désigner les secteurs qui feront l'objet d'un affichage obligatoire.

n° 767 tend à introduire une asymétrie entre les secteurs concernés par l'affichage environnemental.

impose à certains metteurs sur le marché la mise à disposition en des données prises en compte dans l'affichage environnemental, dans une optique de transparence. Le périmètre des données couvertes crée un risque non négligeable de divulgation de données sensibles aux entreprises concurrentes.

À cette problématique de concurrence s'ajoute également le principe de nouvelles contraintes que le législateur juge lui-même excessives pour les petits opérateurs. L'alinéa 10 du présent article ne donne pas d'indication sur la taille des entreprises assujetties à cette obligation, mais il renvoie cet arbitrage au décret d'application. La double incertitude sur le périmètre des données à renseigner et sur celui des entreprises assujetties empêche toute visibilité pour les entreprises.

Billon. Cette disposition, dont la visée est de rendre disponibles les données d'affichage environnemental en lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie, manque de précision quant à l'objectif visé et ne permet pas de garantir la sécurité juridique et le secret industriel nécessaires aux entreprises, comme vient de le dire Catherine Dumas. En effet, la notion de « motif d'intérêt général » n'est pas définie. Si cette notion n'est pas précisée, il convient de limiter à des personnes publiques identifiées la possibilité d'invoquer ce motif. Ces personnes publiques seront destinataires des données, et auront, au préalable, demandé aux acteurs privés concernés le partage desdites données, afin de répondre à une finalité d'intérêt général, qui devra également être précisée. Pour des raisons de sécurité juridique, cet amendement tend à prévoir que les personnes destinataires de ces données soient les administrations rattachées aux ministères de l'économie et de l'écologie. Enfin, les données concernées par la mesure sont précisées pour préserver le respect du droit des affaires et de la propriété industrielle ; le présent amendement vise ainsi à restreindre ces données à celles qui sont affichées en application du présent article.

Il nous semble en effet indispensable de prévoir, d'ores et déjà, cette possibilité de dérive dans la loi. Il s'agit de s'assurer que certains opérateurs économiques ne puissent pas induire le consommateur en erreur en présentant leur propre affichage environnemental, sans garantir l'objectivité des critères retenus pour l'élaborer. En effet, si, pour contrer un affichage qui peut leur être défavorable, certains opérateurs en venaient à développer leur propre affichage avec leurs propres critères, cela aboutirait à une multiplication d'informations, parfois contradictoires, pouvant perdre totalement le consommateur et déboucher sur un dispositif globalement inefficient. Par ailleurs, même en occultant cette volonté d'induire un consommateur en erreur, si un affichage environnemental venait à ne pas remplir l'ensemble des critères fixés dans la loi et le futur décret, il paraîtrait nécessaire de pouvoir l'interdire. Tel est l'objet de cet amendement.

dont le but est de tester des méthodologies et des modalités d'affichage des impacts environnementaux, dans des conditions qui demeurent à déterminer. Par ailleurs, toute information ou allégation environnementale demeure soumise au respect des règles européennes et nationales en

Par ailleurs, plus les délais sont longs pour mettre en oeuvre une mesure et plus les possibilités que celle-ci soit remise en cause ou édulcorée par un autre texte de loi sont fortes. La preuve par l'exemple, avec cet article 1, qui modifie une expérimentation introduite par la loi AGEC du 10 février 2020, laquelle se voit déjà modifiée, un an à peine après sa publication. Les auteurs de cet amendement souhaitent donc réduire ce délai et proposent de le fixer à dix-huit mois, comme dans la loi AGEC et conformément à la demande de la Convention citoyenne pour le climat.

doit entrer en vigueur par décret soit cinq années après la phase d'expérimentation, soit au mieux en 2026. Nous considérons que ce laps de temps est bien trop long et nous proposons de le ramener à deux ans. L'amendement n° 1386, M. Joël Bigot. Cet amendement de repli vise à réduire le temps de la phase d'expérimentation de l'affichage environnemental de cinq à trois ans. Si ce délai n'est pas conforme à la demande de la Convention citoyenne pour le climat, ce que nous regrettons fortement, il représente toutefois un compromis permettant d'envisager la généralisation de cet affichage dans une temporalité plus proche.

de cet article. Je rappelle, par ailleurs, que les cinq ans d'expérimentation sont un maximum ! Dès lors qu'un secteur sera prêt pour une généralisation obligatoire, un décret pourra rendre l'affichage obligatoire plus rapidement. Ces cinq ans d'expérimentation nous donnent une fenêtre de tir large pour traiter l'ensemble des secteurs et disposer d'un affichage pertinent et adapté à la spécificité de chaque secteur. Il faut laisser cette souplesse, d'autant que nous avons prévu, en commission, une généralisation obligatoire prioritaire pour les cinq secteurs les plus avancés.

est à Mme Annick Billon. Cet amendement vise à préciser le cadrage nécessaire à l'expérimentation pour permettre d'en tirer un bilan partagé par l'ensemble des acteurs de la filière concernée. L'expérimentation devra notamment s'attacher à évaluer le degré d'incertitude des données affichées au regard de l'objectif de comparaison des produits entre eux. La méthodologie de l'analyse du cycle de vie repose sur un certain nombre d'hypothèses et de valeurs génériques, qui entraînent une incertitude sur les valeurs d'impact affichées. L'expérimentation doit également évaluer la cohérence de l'affichage environnemental par rapport aux informations environnementales déjà réglementées, comme l'étiquetage Il est essentiel de ne pas créer un millefeuille d'informations sans cohérence entre elles, qui nuirait à la bonne prise en compte, par les consommateurs, des caractéristiques environnementales lors de leur acte d'achat. Quel

à mettre en oeuvre pour les départements d'outre-mer, car il pourrait avoir un impact sur le prix du produit. Dans l'objectif de respecter la justice sociale, une étude d'impact et de faisabilité dans les territoires ultramarins est nécessaire avant la mise en oeuvre de cette proposition. donc pour objet de préciser la prise en compte des particularités des outre-mer, notamment en matière de structuration des prix lors d'éventuelles adaptations de ces expérimentations. Quel est l'avis de la commission ? La première partie de cet amendement est satisfaite par le texte de la commission ; même dans le silence de la loi, il faudra prévoir des dispositions prenant en compte les spécificités des territoires régis par l'article 73 de la Constitution. La seconde partie pose davantage de difficultés, notamment juridiques. Il me semble délicat de poser, dans le principe de la répartition des coûts occasionnés par l'affichage environnemental. Je pense qu'il faut laisser les distributeurs s'organiser avec la chaîne économique, en amont. Je demande donc le retrait Cet amendement vise à garantir que les expérimentations prendront bien en compte les particularités des territoires ultramarins. Une progressivité importante est prévue pour la mise en oeuvre de l'affichage environnemental afin d'évaluer la faisabilité pour les différentes catégories de produits, au travers d'une phase expérimentale. Cette phase est ouverte aux entreprises des territoires d'outre-mer, qui peuvent se faire accompagner par les pouvoirs publics. Elles pourront tester différents paramètres, y compris l'impact sur les prix. Lors de l'examen du texte en commission, la mention du besoin d'une attention particulière aux territoires a été ajoutée au texte de l'article 1, ce qui inclut les territoires d'outre-mer. L'amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer,

visant à élaborer un affichage environnemental qui n'auraient pas été validées dans le cadre de ces expérimentations ou pour les produits d'élevage qui reposent sur la seule méthode de l'analyse du cycle de vie.

il faut garantir une équité de traitement des producteurs par rapport aux méthodes d'évaluation retenues. C'est un principe important à respecter. Cet amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur les inquiétudes d'une grande partie du monde de l'élevage

En pratique, un affichage s'appuyant sur l'analyse du cycle de vie pourrait conduire les consommateurs à acheter en priorité des viandes issues des systèmes les plus intensifs

De multiples initiatives d'affichage environnemental fleurissent actuellement. Force est de constater qu'elles sont prématurées au regard de la fiabilité des données disponibles et des méthodologies d'évaluation environnementale, comme en témoigne l'expérimentation prévue par la loi AGEC, qui est d'ailleurs toujours en cours. en cours. L'affichage environnemental a pour objet d'apporter une information compréhensible, harmonisée et fiable aux consommateurs, en s'appuyant sur les résultats d'une évaluation quantitative,

Quel est l'avis de la commission ?

Cet amendement vise à définir les modalités transitoires d'affichage durant les expérimentations, en imposant la mention du caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci. Aujourd'hui, le but est d'encourager le plus grand nombre de filières et d'entreprises à participer à des expérimentations. Il ne me semble donc pas opportun que la loi rende les modalités d'affichage contraignantes durant la phase expérimentale. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

L'alinéa 14 prévoit que l'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement. Si nous partageons cette ambition, nous estimons toutefois que le Gouvernement ne pourra pas faire l'économie d'une analyse globale, à mi-parcours, de l'ensemble des expérimentations en cours. Cette analyse devra s'accompagner de recommandations en vue de lever d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre de l'affichage environnemental et, donc, de faciliter sa généralisation à terme. Ce dispositif vise à s'assurer de la bonne effectivité de la loi en prévoyant un accompagnement accru des différents acteurs qui mettront en oeuvre cet affichage environnemental. ? L'amendement est partiellement satisfait, car l'étude d'impact du projet de loi informe sur le déroulement des expérimentations en cours. Par ailleurs, nous disposons d'autres moyens pour suivre cette question, comme l'audition des ministres, des représentants Bref, nous ne manquons pas de moyens. Il ne me semble donc pas nécessaire de disposer d'un bilan spécifique, sachant que nous votons sur une nouvelle législation sur l'affichage environnemental, qui prend appui sur les enseignements tirés des expérimentations en cours.

En introduisant de tels critères sociaux, nous faisons en sorte que cet affichage environnemental soit un vrai outil et une vraie certification illustrant la volonté de produire de manière durable et raisonnée. Je salue également l'introduction de règles et de critères qui renforcent, avec certitude, la qualité de l'affichage environnemental.

madame la présidente,

en opérant une transposition, du code de l'environnement dans le code de la consommation,

élargie du producteur (REP) l'identifiant unique du producteur. Or les dispositions de l'article 13 de cette loi n'ont pas pour objet de définir des obligations environnementales. Il s'agit en fait de délivrer au consommateur une information claire,

amendement vise à retarder d'un an l'application des contrôles et sanctions prévus à l'article 13 de la loi AGEC, relatif à l'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Afin d'éclairer les consommateurs, cet article prévoit d'établir un cadre général en matière d'informations sur les qualités et caractéristiques environnementales. Nous sommes très favorables à ce dispositif, mais, en raison du contexte sanitaire et de ses conséquences sur les activités de l'ensemble des acteurs économiques, nous proposons simplement de décaler d'une année

ses promoteurs oublient le fait que les pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Il s'agit là de sanctions suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre les pratiques illicites de « franco-lavage

car celui-ci permet de clarifier les règles d'appréciation de l'origine des biens et de sécuriser le dispositif introduit par l'Assemblée nationale, que nous avons réécrit en commission.

Cet amendement vise à rendre plus visibles, pour le consommateur, les conséquences de la production de textiles à base de microfibres plastiques. Sans une telle information, les procédés de fabrication et leurs effets sur l'environnement restent inconnus du consommateur. Cette mention doit donc figurer quelque part, par exemple sur une étiquette cousue sur les produits eux-mêmes, afin que toute personne faisant l'acquisition de tels produits soit consciente des répercussions que leur fabrication a sur l'environnement. Je vais me permettre d'insister

Oui, il faut une bonne et complète information du consommateur, et il faudrait, pour tout textile contenant des fibres microplastiques, une mention selon laquelle la fabrication et l'utilisation de ce produit « relarguent » des microfibres plastiques dans

de la loi AGEC, relatif à l'information des consommateurs au sujet des qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, est en cours de concertation avec les parties prenantes et sera bientôt en consultation publique prévoit justement une information obligatoire des consommateurs sur le fait que les produits textiles, constitués en majorité de fibres synthétiques, occasionnent des rejets de fibres microplastiques. Votre amendement

À cet égard, il me paraît pertinent de garantir que ces plateformes participent également à l'information du consommateur sur les obligations environnementales des différentes parties prenantes. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? ? Cet amendement a pour objet d'étendre au domaine environnemental les obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques qui mettent en relation des consommateurs avec des professionnels ou des non-professionnels, sans autre précision.

sur cet article, car il vise un objectif crucial. En plaçant, au travers de cet article, l'éducation à l'environnement et au développement durable au coeur des enseignements scolaires, on veut faire des citoyens des générations futures de véritables citoyens écoresponsables. Familiariser nos enfants avec les enjeux de l'environnement doit effectivement être au coeur des politiques éducatives. Cet article prévoit que l'éducation à l'environnement sera dispensée tout au long de la formation scolaire. Si l'on ne peut qu'approuver ce principe, il conviendra néanmoins, avant de confier encore de nouvelles missions et prérogatives à nos enseignants, de s'assurer que ceux-ci disposent des moyens suffisants pour assurer ces enseignements dans le temps qui leur est imparti. Il serait également pertinent de créer une matière scientifique multidisciplinaire relative non seulement au développement durable, mais aussi au domaine de l'énergie, du climat et du civisme. Lors de nos travaux en commission, Mme la ministre a déclaré : « Tout commence à l'école de la République. » C'est vrai ! L'éducation à l'environnement ne pourra pas se passer d'une éducation au civisme, car les incivilités représentent un enjeu environnemental déterminant, notamment au travers des dépôts sauvages et des petits gestes du quotidien qui détériorent la qualité des espaces publics, qui contribuent à dégrader notre environnement et qui finissent par perturber l'usage des espaces verts et des lieux publics.

Cette théorie démontre en effet que les petits détails du quotidien et les incivilités répétées suffisent à transformer un quartier paisible en une véritable jungle, qu'il s'agisse de criminalité ou d'atteintes à l'environnement. La gestion des incivilités nécessite une réelle éducation à la civilité. La prévention scolaire représente un vecteur de diffusion et d'appropriation des règles. La conscience écologique d'appartenir à un environnement implique des droits et des devoirs, le droit de disposer d'un environnement sain, mais surtout le devoir de ne pas le polluer.

Folliot, sur l'article. À l'heure où, dans notre société de consommation, les slogans publicitaires racoleurs et l'information du consommateur se côtoient de manière confuse, les citoyens-consommateurs se doivent de savoir décrypter les annonces et propositions qui leur sont faites. trop nombreux à ignorer les conditions générales de vente, trop complexes, qu'ils acceptent pourtant. Ils sont également trop nombreux à se plaindre du manque ou de la trop grande technicité des informations figurant sur les produits qu'ils achètent. Trop de ménages souffrent de surendettement

à l'Assemblée nationale, et qui visait à introduire des cours d'éducation à la consommation dans les programmes des établissements d'enseignement.

Après la réécriture de cet article en commission, le présent amendement vise à réintroduire la notion de transition écologique, qui a

Le développement durable est une notion sur la base de laquelle s'est construite l'éducation aux enjeux environnementaux, si bien qu'elle résume aujourd'hui l'ambition des programmes scolaires sur le sujet. La prise en compte des possibilités de développement des générations futures est en effet une question centrale lorsqu'on aborde les questions environnementales. Néanmoins, si cette terminologie a bien été utile pour sensibiliser les élèves dans leur cursus, pendant de nombreuses années, elle est aujourd'hui insuffisante pour appréhender, dans sa globalité, la crise écologique. L'éducation en la matière doit être à la mesure des enjeux qui se présentent aux nouvelles générations. Son rôle est d'amener les élèves à réfléchir aux problèmes socioécologiques de notre temps, en les abordant dans leur complexité, sans toutefois imposer le développement durable comme unique perspective de réflexion. D'où cet amendement, qui vise à à élargir la portée de l'objectif éducatif du présent article en y intégrant une approche pluridisciplinaire ainsi qu'une vision plus étendue des enjeux environnementaux abordés.

un objectif de sensibilisation et d'éducation à la consommation responsable et équitable, en complément de l'éducation à l'environnement et au développement durable. La consommation responsable et équitable doit être encouragée dès le plus jeune âge, car elle contribue à faire émerger de nouveaux comportements individuels et collectifs. Il s'agit d'une condition indispensable pour changer en profondeur les pratiques de consommation de notre société, en favorisant la compréhension des interactions complexes entre les modes de consommation et les enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, économiques et sanitaires. L'amendement n° 408, de Marco. Cet amendement vise à mettre en place une transdisciplinarité dans l'enseignement des enjeux environnementaux. Ceux-ci sont aujourd'hui abordés séparément dans toutes les disciplines. Or cette pédagogie n'apporte pas de vision globale et cohérente sur le sujet. Je vous propose donc d'adopter cet amendement de décloisonnement de l'enseignement des enjeux environnementaux, afin que la jeunesse soit mieux informée sur le sujet.

Ça tombe bien, [ ...] des professionnels neutres, dont c'est le métier d'étudier ces questions scientifiquement, loin des débats passionnés mais pas toujours rationnels ou étayés qui fleurissent partout, ont des propositions concrètes et démontrent que sur le long terme tout le monde y gagne.

rédigé par Elena Pasquinelli et Gérald Bronner, pour le Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN), il est rappelé que « Notre société est confrontée à des défis majeurs de santé publique, de développement durable et d'information de masse. Afin d'effectuer des choix informés dans ces domaines ou dans d'autres, il est nécessaire d'être capable de distinguer les connaissances [des] opinions, mais aussi de différencier les informations qui méritent notre confiance de celles qui ne présentent pas de garantie suffisante de fiabilité. L'esprit critique y est alors défini comme « la capacité de calibrer correctement la confiance que l'on a dans certaines informations, grâce à un processus d'évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations, en vue de prendre une décision. »

et à l'effondrement de la biodiversité liés aux activités humaines. C'est pourquoi nous proposons d'introduire une notion plus large de transition écologique, plus à même de rendre compte de la complexité des enjeux auprès des élèves et de les sensibiliser à ces sujets très importants. Quel est l'avis de la commission ?

L'amendement n° 1959 rectifié tend à mettre les enjeux sanitaires de l'éducation à l'environnement en première place, ce qui me semble en contradiction avec la rédaction de l'article. Par ailleurs, la formulation proposée n'est pas meilleure que celle qui figure actuellement à l'article 2, car elle fait mention par deux fois du mot « enjeux », ce qui complique et déséquilibre la rédaction de l'alinéa, sans apporter d'élément particulièrement nouveau.

L'amendement n° 1219 rectifié est également satisfait, car l'éducation au développement vise précisément à favoriser une consommation responsable et équitable. La précision n'apporterait donc pas d'élément nouveau dans cet article ; elle conduirait au contraire à compliquer la rédaction, qui doit rester simple dans un objectif de clarté de la loi. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable. L'amendement n° 408 est satisfait, car l'éducation au développement durable se fera bien de manière transdisciplinaire et dans chaque discipline.

permettra d'inscrire l'éducation au développement durable parmi les dispositions générales constituant le socle de l'éducation. Il souligne notamment la transdisciplinarité de cette éducation et la nécessité d'une continuité pédagogique tout au long du parcours scolaire. Je me permets également de souligner

tend paradoxalement à réduire le champ de cette éducation transversale, en cantonnant celle-ci à une approche strictement environnementale. Or l'éducation au développement durable vise tous les champs de la société, tant économiques que sociaux et environnementaux.

Le réchauffement climatique est en effet en tête des préoccupations des jeunes adultes, dans une proportion qui n'a jamais été si importante. Les jeunes ont donc très bien intégré l'idée que le monde sera profondément bouleversé par le dérèglement climatique. En revanche, on constate l'absence de remise en cause du modèle consumériste des jeunes, qui restent encore peu impliqués dans les « écogestes ». La sensibilisation aux enjeux du changement climatique est forte ; elle mobilise les jeunes, mais elle ne suffit pas à changer les comportements. Or la transition bas-carbone implique des évolutions importantes des modes de vie et de consommation. Ces évolutions doivent s'inscrire dans une société qui porte des valeurs différentes et qui rendra acceptables, voire désirables, d'autres modes de vie. Notre amendement a pour objet de compléter l'éducation aux enjeux environnementaux par une sensibilisation à la nécessité d'adopter de nouveaux comportements plus sobres et plus durables, tant individuels que collectifs. l'avis de la commission ? Cet amendement est satisfait, car c'est le but de l'éducation au développement durable que de favoriser des modes de vie plus sobres et durables. Il faut, je le répète, privilégier une rédaction simple, d'autant que votre préoccupation

ont révélé que ce secteur est responsable de 2 % des émissions de gaz à effet de serre, ce chiffre pouvant tripler d'ici à 2040. Le renouvellement fréquent des terminaux n'est pas anodin, puisque la fabrication de ceux-ci représente 70 % de l'empreinte carbone du numérique. Il est donc primordial que chaque citoyen soit, dès le plus jeune âge, conscient des impacts de sa consommation numérique et du cycle de vie des objets qu'il utilise, bref, qu'il soit sensibilisé à la sobriété numérique. C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter l'article 2 relatif à l'éducation à l'environnement et au développement durable, afin de promouvoir, auprès des élèves, l'information sur les pratiques de sobriété numérique. Il s'inscrit dans la lignée de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui recommande d'accompagner l'évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux.

Notre ambition environnementale doit nous pousser à mettre en place des contenus pédagogiques de qualité, pour mieux connaître la richesse de l'environnement qui nous entoure. Aussi, cet amendement vise à inclure la notion de biodiversité aquatique dans le présent article, afin de sensibiliser les élèves aux menaces anthropiques qui pèsent sur les milieux naturels que sont les fleuves, les lacs et les rivières, ainsi que sur toute la variabilité des organismes aquatiques qui les peuplent. Il existe aujourd'hui 200 aires marines éducatives et 100 aires terrestres

Je suis favorable à cette précision, qui permet d'inclure explicitement la biodiversité de l'eau douce, en plus de la biodiversité marine. La commission a donc émis un avis favorable

En tant qu'ancienne secrétaire d'État chargée de la biodiversité et qu'actuelle ministre de la transition écologique, je peux vous le garantir, la biodiversité aquatique est déjà couverte par la rédaction actuelle du texte. En effet, la biodiversité dite « terrestre » inclut bien le vivant des lacs et des cours d'eau, par exemple. Je vous propose donc de retirer votre amendement, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable.

Cet amendement vise à favoriser un comportement responsable et civique des Français des nouvelles générations, afin d'en faire des citoyens en mesure de comprendre les enjeux des débats liés à la préservation de la biodiversité marine et terrestre. Il s'agit de permettre aux jeunes générations d'être plus sensibilisées à l'impact de leurs comportements, par la construction et l'apprentissage d'une citoyenneté environnementale.

Je suis favorable au fait de préciser que la préservation de la biodiversité doit s'appliquer à l'ensemble du territoire national. Avis favorable. Quel est

C'est la base. Pour autant, sur ce sujet comme sur quelques autres, nos territoires ultramarins sont des laboratoires de la République : ils présentent des singularités fortes dans le domaine de l'environnement et du développement durable, au regard notamment des effets du changement climatique

comme constitutive de l'enseignement du développement durable. Il s'agit d'introduire, de façon pérenne, dans le système éducatif les valeurs de l'économie sociale et solidaire, telles que la coopération la poursuite de l'utilité sociale, et de faire connaître aux collégiens et aux lycéens les différentes composantes d'un secteur qui représente une part de plus en plus importante de l'emploi en France. L'objectif est de renforcer la compréhension des enjeux environnementaux mais aussi économiques et sociaux, ces trois notions étant d'ailleurs au coeur de la définition du développement durable. Quel

du présent article, compte tenu de l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, dite Chaize, car ces dispositions y figurent déjà. Quel est l'avis du Gouvernement ?

l'allié du développement durable, notamment parce que les nouvelles technologies, dont les, démultiplient les possibilités d'évaluer et de modéliser les impacts du changement climatique. Ce sujet riche et complexe

L'intérêt pédagogique du dispositif est triple : il a pour ambition de former, dès le plus jeune âge, à l'écocitoyenneté, de redonner, pour les élèves, du sens au lien homme-nature et de permettre à ces derniers d'échanger avec des acteurs de l'environnement.

encadrés par leurs enseignants et par une structure de l'éducation à l'environnement, se réunissent sous forme d'un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative. Il existe aujourd'hui 200 aires marines éducatives et 140 aires forestières éducatives, déployées dans plus de 300 établissements scolaires situés dans l'Hexagone et en outre-mer. Au travers de cet amendement, nous proposons de dynamiser et d'encourager le développement en réseau des 1 000 premières aires éducatives, afin de sensibiliser les générations futures à la préservation de la biodiversité et à l'écocitoyenneté. Quel

: La parole est à Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à affirmer, au sein même du code de l'éducation, le caractère résilient de l'éducation manuelle. En effet, en confrontant les jeunes générations à la notion de durabilité des objets à la réparation, l'éducation manuelle permet de faire naître des pratiques plus résilientes face à la diminution des ressources, afin d'éviter le gâchis et donc la

dans le virtuel. Éduquer et former, c'est permettre à tout enfant de se réaliser, d'être acteur de sa vie, et donc, non seulement de ne pas rester passif, mais de comprendre la valeur des choses parce qu'on les fait soi-même, parce qu'on y passe du temps. Lors de cette pandémie cette pandémie qui a été riche d'enseignements, l'éducation manuelle aurait d'ailleurs été d'un grand secours, ne serait-ce que pour permettre aux enfants de fabriquer des masques. Imaginez comme les enfants auraient pu participer, s'investir dans l'élan de solidarité nationale ! Dans cette situation si difficile à vivre, ils auraient pu être des acteurs impliqués, être reconnus et faire partie de ceux

Cette précision relative au caractère résilient de l'instruction manuelle me paraît mal s'insérer dans l'article L. 111-2 du code de l'éducation, que vous visez, ma chère collègue. Par ailleurs, votre amendement est satisfait, dans son esprit, par la mention explicite des savoir-faire,

Bigot. Cet amendement vise à renforcer l'éducation à la nature des élèves, grâce aux activités périscolaires. Le temps périscolaire est en effet l'occasion de mener des actions de sensibilisation des élèves, en lien avec les collectivités locales, les associations locales et les professionnels responsables de la gestion et de la préservation des espaces verts, des cours d'eau et des forêts. La rencontre d'acteurs locaux et les sorties sur sites sont des évènements marquants dans le parcours des élèves et constituent des outils majeurs d'apprentissage, qu'il est proposé de valoriser et d'inscrire de façon pérenne dans le parcours éducatif. monsieur le rapporteur,

? Cet amendement vise à introduire les activités de découverte de la nature parmi les activités périscolaires déjà mentionnées dans le code de l'éducation. L'article L. 551-1 de ce code évoque actuellement les activités culturelles et sportives, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais non les activités de découverte de la nature. Or le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer, a d'ores et déjà encouragé le déploiement de l'« école dehors notamment ces dernières semaines. Il a également souhaité renouveler, pour le prochain été, le projet innovant, lancé l'été dernier, des « vacances apprenantes ». Vous le savez, cette nouvelle démarche vise à favoriser une certaine continuité pédagogique, avec des dispositifs tels que l'« école ouverte notamment l'« école ouverte buissonnière », ainsi que l'ensemble des dispositifs des « colos apprenantes », associant renforcement des apprentissages et activités de loisir autour de grands thèmes, comme la culture, la citoyenneté, le sport et le développement durable. Je précise d'ailleurs qu'un guide d'activités d'éducation au développement durable avait été rédigé l'an dernier à destination des animateurs et qu'il sera substantiellement enrichi cette année et publié dès la fin de ce mois de juin. Ainsi, votre amendement étant déjà satisfait, je m'en remets

de Marco. Cet amendement vise à prévoir la mise en place d'un plan national de sensibilisation à la transition écologique global et transversal, concernant non seulement l'éducation nationale, mais aussi l'ensemble de la population française. plan permettra notamment de soutenir la diffusion de documentaires ou d'autres campagnes de communication pour sensibiliser enfants et adultes à la transition écologique. Mes chers collègues, la connaissance du problème étant essentielle pour agir, je vous invite à adopter cet amendement. Il ne me semble pas nécessaire de prévoir un tel plan national de sensibilisation à la transition écologique dans la loi. Des campagnes d'information peuvent être organisées pour viser le même objectif, tout à fait louable, sans qu'il soit besoin de formaliser impérativement un plan ayant une existence législative.

Cet amendement vise à prévoir que les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) fixent les objectifs de moyen et long termes des régions en matière de sensibilisation au développement durable. En effet, les régions, en tant que chefs de file sur de nombreux sujets environnementaux, ont un rôle clé à jouer en la matière. Par ailleurs, leurs actions en matière environnementale seront d'autant plus facilitées et reconnues que les citoyens sont sensibilisés et convaincus de l'importance des enjeux. l'avis de la commission ? Cet amendement

? Les Sraddet portent avant tout des objectifs quantitatifs en matière d'environnement et d'aménagement, associés à des orientations et des investissements, en particulier dans les infrastructures. Il me paraît donc assez artificiel d'ajouter une telle attribution aux Sraddet. Par ailleurs, la sensibilisation à l'environnement ne relève pas des régions. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable

Nadège Havet. La sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux, dans le cadre du service national universel (SNU), est une obligation. Les jeunes doivent en effet être sensibilisés et oeuvrer en faveur de l'environnement durant cette phase de cohésion. En outre, la gestion du quotidien au sein du SNU doit être pensée comme une occasion complémentaire de sensibiliser les jeunes aux problématiques environnementales. Les jeunes pourront ensuite poursuivre leur engagement pour l'environnement dans le cadre de la mission d'intérêt général qu'ils réaliseront, voire dans le cadre d'un engagement volontaire dans une association oeuvrant dans le domaine de l'environnement. Cet amendement tend donc à mentionner explicitement la sensibilisation aux enjeux environnementaux et de développement durable parmi les obligations du service national universel, étant entendu que des actions existent d'ores et déjà dans ce cadre. Cette sensibilisation doit permettre de rassembler toute une classe d'âge autour des conséquences des différentes pollutions sur notre écosystème et doit s'articuler autour d'activités pratiques ancrées territorialement. Quel est l'avis de la commission ? dans l'article L. 111-2 du code du service national, qui pose les principes fondamentaux de l'organisation du service national, avec le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement.

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à revenir sur la position de la commission, qui a adopté cet article 3 avec des modifications. Je trouve dommage de supprimer l'ensemble de ces dispositions, alors qu'elles sont nécessaires pour la conduite de la politique éducative nationale et locale. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

une liste d'exemples sera, comme souvent, toujours trop restrictive. Il est indispensable que, dans un cadre national, les chefs d'établissement disposent de la liberté nécessaire pour faire des choix de partenariat adaptés aux spécificités locales, c'est-à-dire à l'environnement non seulement naturel, mais encore institutionnel, social et pédagogique de leurs élèves. Or, si les associations sont effectivement des partenaires privilégiés, au même titre que d'autres acteurs- les collectivités territoriales ou les acteurs de la santé

lutte contre « la violence ». Il est vrai qu'il existe, au sein de l'éducation nationale, un grand nombre de dispositifs visant à mieux protéger les élèves, en identifiant précisément les différents types et origines des violences auxquelles ils peuvent être confrontés. Il y a donc une justification à passer d'un singulier indéfini à un pluriel d'action.

La santé environnementale est au coeur d'une demande citoyenne de lien entre environnement et santé, en complément de l'éducation au développement durable. L'article 1 de la Charte de l'environnement précise bien : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Quel est l'avis de la commission ?

de l'Assemblée nationale. Il tend à réaffirmer que le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est un espace de conception, de dialogue et d'animation de projets relatifs à l'éducation à la sexualité,

Cet amendement tend à rétablir une phrase supprimée par la commission. Pour ma part, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Quel est

En effet, ces associations sont des acteurs dont la connaissance et le respect des espaces naturels, de la faune et des enjeux liés au développement durable résultent d'une expérience concrète des réalités du terrain. À ce titre, elles

L'impact des déchets sur l'environnement représente un enjeu considérable ; 81 000 tonnes de déchets sauvages sont rejetées dans la nature, chaque année,

Cet amendement vise donc à instaurer une journée nationale de l'environnement, fixée au 5 juin, date à laquelle se déroule également la journée mondiale de l'environnement. Cette journée nationale sera l'occasion de sensibiliser les jeunes générations à cette problématique, en favorisant l'organisation d'actions éducatives. Quel est

D'un autre côté, une journée nationale permettrait d'afficher une priorité politique forte. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat. Quel est